Monsieur le président, La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée,

Monsieur le président, monsieur le président de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le texte aujourd'hui soumis à votre approbation est l'aboutissement d'un long travail, dont l'impulsion a été donnée par le Président de la République lors de son discours prononcé à Ouagadougou en novembre 2017 il y avait exprimé sa volonté de réunir les conditions nécessaires à des restitutions d'oeuvres relevant du patrimoine africain, dans le cadre du renouvellement et de l'approfondissement du partenariat entre la France et les pays du continent africain. C'est un texte important, qui ouvre une nouvelle page dans nos relations culturelles avec le continent africain. Il n'est pas question ici de repentance ou de réparation. C'est l'avenir qui nous intéresse, et il passe par la refondation du lien culturel qui unit la France à l'Afrique. S'il est inédit par son ampleur et sa symbolique, le projet de restitution des vingt-six oeuvres issues du « Trésor de Béhanzin » à la République du Bénin, que du sabre attribué à El Hadj Omar Tall et de son fourreau à la République du Sénégal, s'inscrit néanmoins dans le prolongement d'une politique de coopération culturelle déjà engagée avec ces deux pays. Ce projet de loi s'inscrit également dans un contexte de réflexion sur le rôle et les missions des musées en Europe et dans le monde. Le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy remis au Président de la République en 2018 a été l'occasion de passionnants échanges sur l'histoire des collections, notamment originaires du continent africain, et sur la nécessité de mieux en expliquer la provenance au grand public. Les oeuvres et les objets que nous souhaitons restituer au Bénin et au Sénégal sont exceptionnels à tous égards. Témoins d'un passé glorieux et tourmenté, leurs qualités esthétiques attestent le génie de leurs créateurs et leur valeur symbolique n'a cessé de s'accroître au cours du temps. Ils sont devenus de véritables « lieux de mémoire », au sens que l'historien Pierre Nora donne à cette expression, dépositaires d'une partie de l'identité des peuples sénégalais et béninois. Le sabre attribué à El Hadj Omar Tall ainsi que son fourreau renvoient, dans l'imaginaire collectif, à la formidable épopée de la fondation et de l'extension de l'empire toucouleur, sous la conduite de ce chef militaire et religieux d'exception, qui a fini par se heurter aux forces françaises. Données au musée de l'Armée il y a plus d'un siècle par le général Louis Archinard, ces deux pièces sont actuellement exposées au musée des civilisations noires de Dakar dans le cadre d'une convention de prêt de longue durée. Les oeuvres du trésor des rois d'Abomey, quant à elles, constituaient la manifestation insigne de la continuité et de la grandeur de cette dynastie pluriséculaire, avant que le général Dodds ne s'en empare, par la force, en 1892. pièces sont les derniers témoins de l'esprit de résistance du roi Béhanzin, qui a préféré incendier son palais et les inestimables qu'il contenait plutôt que de les abandonner aux mains des troupes françaises victorieuses. La perte de ce trésor royal est progressivement devenue, pour le peuple béninois, le symbole d'une indépendance perdue. Conservées par différents musées français puis, à partir de sa création en 1999, par le musée du quai Branly-Jacques Chirac, ces oeuvres ont suscité une émotion considérable lorsqu'elles ont été présentées sur le sol béninois, dans le cadre d'une exposition temporaire. La République du Bénin a, en 2016, demandé à la République française de lui restituer les vingt-six oeuvres du trésor royal d'Abomey. En restituant ces objets d'exception au Bénin comme au Sénégal, nous donnerons à la jeunesse africaine accès à des éléments majeurs de son propre patrimoine et de son identité, conformément au souhait exprimé par le Président de la République. Je souhaite à présent vous préciser le sens, la portée et les conséquences du texte qui vous est soumis. Tout d'abord, il convient de rappeler que cette restitution de biens culturels par un État à un autre État n'a en soi rien d'inédit. Ce qui l'est davantage, c'est- je viens de le souligner -la qualité et la dimension symbolique des oeuvres concernées pour le patrimoine africain comme pour le patrimoine mondial. Parmi les restitutions récentes consenties par la France figurent notamment

Ces différents cas de figure illustrent la diversité des voies offertes par le droit français pour procéder à des restitutions. Dans le cas présent, en l'absence de recours judiciaire du Bénin et du Sénégal, le législateur peut apporter une réponse aux demandes de ces deux pays sans craindre les effets d'une jurisprudence que la décision du juge aurait nécessairement fait naître. Sans portée générale, ce projet de loi ne vaut que pour le cas spécifique de l'ensemble des objets qu'il énumère expressément. Il n'institue aucun « droit général à la restitution », en fonction de critères abstraits qui seraient définis. La voie La voie législative s'impose à nous, par ailleurs, dans la mesure où la restitution des objets au Bénin et au Sénégal implique de déroger au principe d'inaliénabilité des collections publiques, inscrit dans le code du patrimoine. Mais si ce projet de loi tend à contrevenir ponctuellement à ce principe, il ne le remet nullement en cause, pas plus que ne l'ont fait les lois précédentes du même type, comme celle de 2010. l'amendement de la députée Constance Le Grip lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale permet d'ailleurs de lever toute incertitude à cet égard, en inscrivant dans le texte la référence à ce principe et en désignant explicitement ces restitutions comme des dérogations. À l'inverse, l'amendement adopté par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, ajoutant au projet de loi un article 3 instaurant un « Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d'oeuvres d'art extra-occidentales me semble nous éloigner, au profit d'un dispositif-cadre, de cette logique « d'espèce », cette appréciation au cas par cas que le Gouvernement privilégie pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est pourquoi j'en proposerai la suppression. Au-delà des points juridiques, ces restitutions soulèvent des questions purement politiques, au sens le plus noble du mot, sur lesquelles je voudrais apporter un éclairage. Le présent projet de loi n'est en aucun cas une remise en cause ou une critique du rôle joué par les institutions françaises qui ont assuré la conservation de ces oeuvres depuis de nombreuses années, à savoir le musée du quai Branly-Jacques Chirac et le musée de l'Armée- tout au contraire.

Elles en ont également assuré la présentation au public, tant en France qu'à l'étranger, en particulier dans leurs pays d'origine, aujourd'hui concernés par ces restitutions, sous la forme de prêts. Nous devons leur en être reconnaissants. Accepter ces restitutions, ce n'est pas davantage remettre en cause le modèle universaliste de nos musées, que nous devons plus que jamais défendre. Le contexte actuel, dans notre pays comme à l'étranger, nous rappelle de la façon la plus tragique à quelles extrémités monstrueuses les crispations identitaires et le mépris de la culture de l'autre peuvent conduire. La mission de la France, aujourd'hui plus encore qu'hier, est de favoriser, notamment grâce à la circulation des oeuvres, le dialogue des cultures et l'échange des perceptions. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je veux vous le dire ce soir avec gravité la fonction première de la culture est d'exprimer et d'explorer ce que notre condition humaine a d'universel. Cette conviction, qui est au fondement de notre ministère français de la culture, peut paraître aujourd'hui, hélas, de moins en moins partagée. Ce projet de loi est aussi une façon de rappeler que nous n'y renoncerons jamais. C'est au nom d'une telle conviction, d'un tel idéal, que la France n'accepte de restituer des oeuvres à d'autres États que si ces États s'engagent à ce que ces oeuvres gardent leur vocation patrimoniale, c'est-à-dire continuent à être conservées et présentées au public dans des lieux consacrés à cette fonction. Dans le cas du Bénin et du Sénégal, ces garanties ont été données. La France accompagne les initiatives de ces deux pays en faveur du patrimoine, bien au-delà des seules restitutions. est le sens du programme de travail commun élaboré avec le Bénin ainsi que du partenariat culturel renforcé avec le Sénégal, qui visent tous deux à inscrire ces restitutions dans le cadre plus large d'une véritable coopération ambitieuse. Nous soutenons ainsi des projets de développement de musées et des actions de formation, qui permettront de partager l'expertise des professionnels français du patrimoine et de mettre en place de véritables filières professionnelles dans ce domaine. Le patrimoine d'exception ainsi rendu sera de la sorte accessible, sur le long terme, au plus grand nombre, dans un cadre à la hauteur de sa valeur. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis n'est pas un acte de repentance- je le disais - ni une condamnation du modèle culturel français. C'est un acte d'amitié et de confiance envers le Bénin et le Sénégal, pays auxquels nous lient une longue histoire commune et des projets communs d'avenir. Ce projet de loi permettra aux Béninois et aux Sénégalais de renouer plus directement avec leur passé et d'accéder à des éléments constitutifs de leur histoire, comme nos propres collections nous permettent de le faire. Ces objets symboliques leur permettront de penser un présent et de bâtir un futur qui leur soient propres, tout en faisant l'objet d'un partage avec les autres, avec tous ceux qui visiteront ces nouveaux musées. C'est, pour la France, un honneur et une fierté de pouvoir jouer un rôle actif en la matière, et de contribuer à ce que notre histoire commune, riche sans jamais avoir été simple, ne cesse de nous nourrir les uns les autres et de nous amener à nous dépasser. La parole

visant à contribuer au désir de la jeunesse africaine de connaître et de s'approprier son histoire ? Comment ne pas être favorable à l'objectif de renforcer notre dialogue avec l'Afrique, ce continent ami, par le biais d'une coopération culturelle et patrimoniale accrue ? Ce n'est en tout cas pas le Sénat qui pourrait contester ces deux points, lui qui a été à l'initiative tant des deux seules lois de restitution que notre pays ait jamais adoptées que de la consécration législative des droits culturels.

les revendications du Bénin et du Sénégal portent sur des objets précis et limités en nombre, des biens qui revêtent pour eux une portée culturelle, symbolique et spirituelle, au-delà de la simple valeur artistique et historique qu'ils ont aussi en France.

visant à faciliter l'accès de leurs populations à leur patrimoine. À cet égard- cet élément était pour nous essentiel -, des garanties ont été données quant aux modalités de conservation et de présentation au public de ces biens au cas où nous acceptions leur cession. Le problème soulevé par ce projet de loi ne tient donc pas à sa démarche. Celle-ci est fondée d'un point de vue éthique et diplomatique ; elle témoigne de la volonté de la France de renouer avec l'esprit des Lumières et, non pas de se repentir, mais de se réapproprier conjointement, dans un cas avec le Bénin, dans l'autre avec le Sénégal, une part importante de notre histoire commune, cette réappropriation devant servir de base à une coopération culturelle renouvelée. Notre pays ne peut en sortir que grandi. Ce qui est en cause, c'est la méthode qui préside à la politique menée en matière de restitution depuis le discours de Ouagadougou, dont ce projet de loi est l'un des volets. Certains pourront trouver ce sujet anodin, mais il y va de collections nationales, c'est-à-dire de biens qui appartiennent au patrimoine de la Nation et qui, à ce titre, sont protégés par le principe d'inaliénabilité, au même titre que le reste du domaine public. C'est ce qui rend indispensable l'autorisation de la représentation nationale pour faire sortir des biens des collections publiques. par le passé, adopté deux lois de restitution, mais le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui s'en distingue à la fois par la forme, puisqu'il s'agit d'une initiative gouvernementale et non parlementaire, et par le fond, dans la mesure où ce texte concerne le retour d'oeuvres et d'objets, et non de restes humains, ces deux types de biens culturels ne pouvant pas être traités de la même manière. Là où la loi de 2010 de restitution des têtes maories avait été précédée d'un vaste symposium international consacré à la question des restes humains dans les musées, organisé au musée du quai Branly en février 2008 à la demande de la ministre de la culture de l'époque, Christine Albanel,

associé les scientifiques à leurs travaux pèse pour beaucoup dans les critiques dont leur rapport fait l'objet. Il est vrai que les conservateurs des musées concernés ont été consultés pour préparer ce projet de loi ; mais ont-ils pu être véritablement entendus, sachant que le Président de la République avait déjà annoncé publiquement le retour de ces objets ? Le problème, dans cette affaire, est que la décision politique a précédé et prévalu sur toute autre forme de débat, historique, juridique, scientifique, philosophique, au mépris du principe d'inaliénabilité des collections, pourtant instauré pour empêcher le « fait du prince ». Ainsi le débat au Parlement est-il faussé et s'apparente-t-il davantage au vote d'un projet de loi de ratification, dans la mesure où l'État a déjà engagé sa parole et où le sabre a déjà été, il y a un an, officiellement remis au Sénégal- je le regrette. J'en veux pour preuve, aussi, le manque de considération

C'est la même ambition qui a, une fois encore, animé notre commission. Le texte que nous avons adopté la semaine dernière n'a nullement remis en cause le principe du retour des objets. Aucun amendement n'avait même été déposé en ce sens. En revanche, nous jugeons indispensable de garantir, dans le futur, un surcroît de méthode, celle-ci ayant partiellement fait défaut cette fois-ci. Nous sentons tous que l'enjeu de ce projet de loi va au-delà de son simple objet. Certains seront déçus qu'il n'ait pas été l'occasion de poser un cadre général ; d'autres, au contraire, craignent l'effet d'entraînement qu'il pourrait avoir. Ces points de vue contradictoires révèlent toute la complexité du sujet. Ils démontrent aussi combien nous sommes conscients de l'ampleur que sont appelées à prendre les questions de restitution dans les années à venir, eu égard aux revendications toujours plus nombreuses que l'on observe dans le cadre de l'Unesco ou d'autres enceintes internationales. En même temps, nos débats en commission ont révélé notre profond attachement au principe d'inaliénabilité des collections, véritable « colonne vertébrale » de nos musées. D'où la nécessité de définir une procédure qui permette à la fois de préserver ce principe et d'engager un nécessaire travail approfondi de connaissance des oeuvres de nos collections, propre à les mettre en lumière dans toute la vérité de leur histoire. Il s'agit de combler le retard accumulé par notre pays en la matière et de lui permettre de sortir de son isolement.

À nos yeux, la création d'un conseil national de réflexion sur le sujet permettrait de répondre à ce double enjeu. Consulté sur les demandes de restitution présentées par des États étrangers avant qu'une réponse officielle y soit apportée, il permettrait, premièrement, de garantir qu'un temps soit réservé à l'examen scientifique des demandes, avant toute intervention politique et diplomatique. Le conseil agirait comme une protection face au risque que les intérêts politiques et activistes prennent le dessus sur toute autre forme de considération.

en revanche garantir la formation progressive d'une doctrine scientifique en matière de restitution, susceptible de mettre un frein aux demandes tous azimuts. Sa mission ne pourra ainsi se résumer à observer s'il existe un intérêt public attaché à la conservation d'un bien dans les collections ; il s'agira plutôt de mettre en balance cet intérêt public

celui de la recherche et les scientifiques à engager vraiment, cette fois, une réflexion en matière de gestion éthique des collections et de permettre aux autorités françaises de reprendre la main sur le débat relatif aux restitutions. Il est indispensable de clarifier la position française, tant celle-ci est aujourd'hui brouillée par le rapport Sarr-Savoy, qui constitue à ce stade le seul document de référence que brandissent les États étrangers. Je regrette que nous ayons perdu dix ans, car toutes ces missions auraient pu être menées à bien par la Commission scientifique nationale des collections (CSNC) si l'intention exprimée à l'unanimité par le législateur en 2010 avait été fidèlement et correctement traduite. Le Gouvernement a fait le choix de supprimer cette commission, en se gardant bien d'expliquer les raisons à l'origine de ses dysfonctionnements. Dont acte ; nous en tirons les leçons, et aussi le bilan- car bilan il y a ; nous aurons l'occasion d'en reparler la création de ce conseil national- le mot « conseil » est essentiel -spécifiquement consacré aux questions de restitution et de réflexion sur les collections. Vous le voyez, madame la ministre : le Sénat attache beaucoup d'importance à ces questions de circulation et de retour des oeuvres lorsque cela apparaît justifié. Il est soucieux, pour autant, de l'authenticité et de la rigueur de la démarche C'est la raison pour laquelle notre commission est attachée à la création de cet outil garantissant une pérennité de la réflexion bien au-delà des gouvernements qui passent

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme / Qui s'attache à notre âme et l'oblige d'aimer ? » Ces vers de Lamartine illustrent parfaitement la charge affective pesant, pour des individus ou tout un peuple, Qu'est-ce qui arrache un objet à sa banalité pour le hisser au rang d'oeuvre d'art ou de bien culturel ? Ce peut être sa dimension esthétique, sa matière, son origine, son secret de fabrication ou simplement son parcours historique l'ayant fait passer dans les mains de telle ou telle personne illustre. Nous ne pouvons nier l'apport culturel de l'art africain dans l'élaboration de notre propre culture. Il a permis en retour de repérer, et parfois de sauver de la destruction, du vol ou du trafic, certains biens africains, leur conférant ainsi une dimension culturelle qu'ils n'auraient pas eue. Ce retour participe au rayonnement universel de la culture française. Ce projet de loi concrétise un engagement fort du Président de la République formulé au Burkina Faso en novembre 2017 devant les étudiants de l'université de Ouagadougou : restituer à l'Afrique des biens culturels appartenant à son patrimoine. Cette démarche s'inscrit plus largement dans le cadre d'une refondation des relations avec nos homologues africains. La coopération culturelle en est un des piliers majeurs. Il s'agit de permettre aux peuples africains d'avoir accès, chez eux, aux oeuvres issues de leurs propres cultures et de leur civilisation, alors que 90 % de leur patrimoine se situe aujourd'hui hors du continent africain, essentiellement dans les musées européens. Cette nouvelle impulsion démontre la volonté de la France d'établir une amitié renouvelée avec ses partenaires africains. Ce projet de loi vise, en outre, à mettre le droit français en conformité avec une politique de restitution réfléchie dans cette perspective. Il entend également autoriser une dérogation limitée au principe général d'inaliénabilité applicable aux collections publiques françaises, afin de laisser sortir ces objets des collections nationales dans le cadre d'un transfert de propriété. Cette démarche mérite d'être éclairée par un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d'oeuvres d'art extra-européennes. Les précédents Les précédents notables ont participé à l'affermissement de nos relations bilatérales, à l'instar des restitutions de la dépouille mortelle de la Vénus hottentote à l'Afrique du Sud en 2002 ou du transfert des têtes maories à la Nouvelle-Zélande en 2010. Pour autant, ce projet ne vise pas à remettre en question ce principe d'inaliénabilité, ni même la vocation universaliste des musées français. Il ne s'agit pas de vider nos collections ; ces restitutions sont limitées à certaines oeuvres et doivent le rester. Elles répondent à des demandes précises des pays, et s'effectuent avec des garanties de bonne conservation. En effet, le Sénégal et le Bénin bénéficient d'ores et déjà d'une solide expertise et d'une volonté forte de valoriser leurs collections. De plus, ces retours sont porteurs d'un message fort à destination de nos homologues africains. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de diplomatie culturelle. Ce geste doit permettre de tourner la page de la Françafrique et participer à la construction d'un nouvel imaginaire, loin des souvenirs de nos conflits et de nos traumatismes. En effet, nous restituons des objets soustraits à leurs pays d'origine sous la colonisation en l'absence de cadre juridique légal. Il est nécessaire de prendre conscience des enjeux mémoriels et d'accéder aux demandes légitimes des peuples africains de reconnexion avec leur patrimoine. Car ces oeuvres sont empreintes d'une forte charge symbolique, spirituelle et historique. oeuvres du trésor royal d'Abomey, conservées par le musée du quai Branly-Jacques Chirac à la suite de leur don aux collections nationales par le général Alfred Dodds, seront restituées au Bénin. Elles constitueront les pièces maîtresses du futur complexe muséal d'Abomey, conçu en étroite collaboration avec l'Agence française de développement (AFD), qui viendra renforcer le développement touristique local. Le sabre dit d'El Hadj Omar Tall, conservé par le musée de l'armée à la suite d'un don du général Louis Archinard, sera restitué au Sénégal. au Sénégal. Actuellement prêté au musée des civilisations noires de Dakar, il en constitue déjà une des oeuvres majeures. Enfin, il s'agit d'un acte de confiance à destination de la jeunesse africaine, alors que 70 % de la population a moins de 30 ans. La France sera au rendez-vous pour aider le continent à relever les défis contemporains. Elle l'aidera ainsi à se réapproprier son histoire et à mettre fin à une forme de captation patrimoniale. Les retours de biens culturels doivent ainsi s'intégrer dans une coopération patrimoniale et muséale étendue. Celle-ci pourrait passer par le déploiement de l'expertise de l'Agence France-Museums dans les pays africains ou le renforcement de la formation de leurs conservateurs et de leurs restaurateurs d'oeuvres d'art. Ce travail devra trouver un équilibre entre l'exigence de préservation du patrimoine présent dans les musées français et une circulation renforcée des oeuvres par l'intermédiaire de restitutions, de retours ou de prêts,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le 9 thermidor de l'an VI de la République, sur le Champ de Mars à Paris, s'ébranla le long convoi des oeuvres d'art spoliées par Napoléon lors de sa campagne d'Italie. Dans l'un des nombreux charriots se trouvaient les chevaux de cuivre de la basilique Saint-Marc de Venise. Ces statues auraient été fondues au IV siècle avant notre ère, dans une île grecque du Dodécanèse, puis installées sur la de l'hippodrome de Constantinople et, enfin, disposées, en 1204, par les Vénitiens, sur la porte principale de la basilique Saint-Marc. Après leur transport à Paris, Napoléon les plaça au sommet de l'arc de triomphe du Carrousel, mais elles furent rendues à Venise par l'Autriche après la chute de l'Empire. Avec elles, les chars transportaient aussi plus de cinq cents tableaux de maîtres. La moitié d'entre eux fut restituée, mais l'autre resta en France pour constituer le coeur des collections du Louvre. Ainsi va la vie des oeuvres, qui passent de main en main et de pays en pays au gré du pouvoir des princes, de la fortune de la guerre et des alliances des États. Celles qui font l'objet du présent projet de loi auraient pu s'inscrire dans cette histoire tumultueuse, mais les circonstances particulières de la conquête militaire de l'Afrique de l'Ouest font de cette restitution une péripétie supplémentaire de notre relation complexe avec notre histoire coloniale. Par ailleurs, le choix de ces biens culturels, les formes de l'instruction des demandes par les services du ministère de la culture et du musée de l'Armée, les conditions de leur transport et de leur présentation au Bénin et au Sénégal posent de nombreuses questions. Enfin, nous ne comprenons pas comment ces dossiers ont pu, au plus haut niveau, être gérés dans l'ignorance presque totale de l'expérience acquise lors de la restitution des têtes maories et des initiatives fortes défendues par notre collègue la sénatrice Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture du Sénat. Le 25 septembre 2007, à cette même tribune, à l'occasion du débat sur les accords passés entre la France et les Émirats arabes unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi,

le Louvre Abou Dabi constitue un formidable vecteur de rayonnement de l'universalité de la culture et un défi que la France, au nom de la diversité culturelle et du rapprochement des civilisations, se devait de relever. Dans ce cadre, les musées français ont apporté leur expertise en matière de conception du bâtiment, de gestion des collections et prêté trois cents oeuvres. La réussite actuelle de cette institution doit beaucoup à cet investissement majeur et à la qualité du partenariat entre les deux pays. Il est vrai que cet échange a été accompagné par une généreuse participation des Émirats arabes unis de presque un milliard d'euros. L'humanisme n'a pas de prix Le 28 novembre 2017, devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait rappelé que, pour lui, « les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire ce constat, il concluait à la nécessité de renouveler le dialogue franco-africain pas la construction d'un projet commun. Il considérait, à raison, que la culture devait en constituer un chapitre essentiel et souhaitait que les restitutions du patrimoine africain s'organisassent rapidement dans ce cadre. La forme juridique adaptée de ce partenariat aurait dû être, à l'imitation des accords pour le Louvre d'Abou Dabi, un traité international. Le Conseil d'État, dans son avis, a considéré que, dans le cadre de l'article 53 de la Constitution, le transfert de propriété aurait pu être organisé par un accord international. Ce traité aurait eu l'avantage de préciser les engagements de la France, au titre de l'aide au développement, pour le financement du transport des oeuvres, la construction des installations qui vont les accueillir et l'instauration des échanges indispensables entre les institutions patrimoniales des pays. Il aurait pu aussi organiser le prêt aux musées africains d'oeuvres symboliques du patrimoine français. Défendre l'universalité de l'art exige de notre pays des actions volontaires afin de faciliter la circulation des oeuvres par un double processus de reconnaissance. Aimé Césaire disait : « Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'" universel ". Ma conception de l'universel est celle d'un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers. » Je regrette vivement que les présentes restitutions n'aient pas porté cette double ambition. La parole

La question de la restitution des biens culturels y a régulièrement été évoquée par mes interlocuteurs, notamment par Marie-Cécile Zinsou, qui a d'ailleurs été entendue dans le cadre de nos travaux préparatoires. Si ces restitutions font suite à la volonté du Président de la République d'oeuvrer au retour du patrimoine africain en Afrique et à son discours prononcé à Ouagadougou en 2017, elles trouvent également leur origine dans la volonté des États africains de voir revenir sur leur sol les biens culturels dont ils ont été dépossédés pendant la colonisation. Cette demande est fortement appuyée par la société civile africaine et par de nombreuses associations. Ce projet de loi, au-delà du discours du Président de la République, est la réponse à une demande ancienne et forte dont je regrette qu'elle n'ait pas été entendue plus tôt. Précisons d'emblée que cette demande ne concerne pas tous les biens culturels issus du patrimoine africain présents sur notre territoire, notamment au quai Branly,

qui ont été saisis en 1892 par le général Dodds, commandant des armées coloniales françaises, dans le cadre de la guerre du Dahomey, et du sabre attribué à El Hadj Omar Tall, qui aurait été confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893. Cette demande limitée n'est donc pas de nature à remettre en cause le caractère inaliénable des collections auquel nous sommes tous attachés. L'Afrique est un continent jeune- on considère que 19 ans y est aujourd'hui l'âge médian -, qui connaîtra, dans les décennies à venir, une croissance démographique spectaculaire. Ces restitutions peuvent jouer un rôle majeur pour permettre à cette jeunesse de retisser le lien avec son histoire et de renforcer son identité. Pour que ces futures générations construisent leur avenir, il est vital qu'elles puissent accéder à leur histoire et s'inspirer des générations précédentes. Car, comme le disait justement Aimé Césaire, « un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». n'oublions pas les enjeux de mémoire qui se jouent également ici et qui sont vitaux dans la construction et l'avenir de nos sociétés. Dans les discussions que j'ai pu avoir lors de mes déplacements en Afrique, il était souvent question de fierté ou de dignité retrouvée lorsqu'était évoqué le retour de biens culturels sur le sol africain. Ces restitutions sont également rendues nécessaire par le fait que les collaborations, dépôts ou prêts entre musées, bien que précieux, ne sont aujourd'hui pas toujours suffisants, car ils ne répondent plus aux demandes de la société africaine.

avait attiré 275 000 personnes en trois mois, et nombre de Béninois n'avaient pas compris pourquoi les objets de leur patrimoine devaient retourner en France à la fin de l'exposition.

Tall offre ainsi la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre de notre diplomatie culturelle avec l'Afrique. À l'inverse, une fin de non-recevoir aurait des conséquences désastreuses et nuirait fortement aux relations franco-africaines. Les inquiétudes que l'on peut entendre concernant la conservation et la présentation au public de ces biens seront, je n'en doute pas, levées grâce au renforcement de la coopération culturelle franco-béninoise, à la coopération muséale, à la formation de conservateurs de musée, à l'échange d'experts et à un programme de travail commun. Il convient de tout entreprendre pour que ces biens continuent, à l'avenir, d'être présentés au public dans des lieux adaptés.

qui étaient jusqu'à présent exposés dans nos musées sont restitués à des pays africains. Je crains que, sans explication et sans démarche historique accompagnant ces restitutions, ces dernières puissent être mal comprises par notre population fortement attachée à l'histoire et aux enjeux qu'elle peut représenter. En conclusion, ce projet de loi, qui est un geste fort et symbolique, mais de portée limitée sur le plan législatif, pose naturellement la question de l'après. N'en doutons pas, mes chers collègues, d'autres États africains souhaiteront à l'avenir récupérer des biens culturels appartenant à leur histoire.

La question des restitutions a mis au premier plan celle des provenances, un questionnement prégnant dans notre siècle, mais qui ne l'était pas dans le précédent

adopter à l'avenir ? Devrons-nous, chaque fois, passer par un dispositif dérogatoire au droit commun ou, à l'inverse, disposerons-nous d'une loi-cadre qui permettrait, peut-être, une procédure plus claire et plus lisible et dans laquelle pourrait être indiqué que seuls des objets acquis par la violence et la contrainte peuvent être concernés par une éventuelle restitution. La parole

tout d'abord d'avoir une pensée amicale pour notre ancien collègue Alain Schmitz qui s'était impliqué, avec l'intelligence fine qu'on lui connaît, dans cette complexe question des restitutions.

Avec raison, elle appelle depuis longtemps à fixer une méthode là où prévaut, jusqu'à ce jour, une approche trop strictement politique répondant aux seules exigences des relations diplomatiques du moment. Sur un dossier de cette nature, il aurait été bien utile que Catherine Morin-Desailly soit davantage entendue et que le Gouvernement esquisse une méthode fondée sur quelques principes. eux serait d'appréhender la question en se départant d'une approche exclusivement morale, fondée sur une vision du bien et du mal dont on sait qu'elle est variable avec le temps et les peuples.

Mais il aurait également pu être vu comme le retour des symboles de l'oppression de l'ethnie fon sur ses esclaves yorubas, après la chute et le pillage de Kétou en 1886. Je ne suis pas certain que les descendants des Yorubas soient si heureux que cela de les voir réinstaller dans le palais de leurs anciens maîtres. « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà.

Cela aurait évité, dans l'affaire qui nous préoccupe, d'attribuer à un sabre une valeur et une symbolique qu'il n'a peut-être pas et à celui qui est censé l'avoir porté, une aura qu'il ne mérite certainement pas. Les travaux de Francis Simonis ou Bertrand Goy sur le sabre d'El Hadj Omar Tall n'ont-ils pas montré que la légende de ce sabre fut surtout forgée par le général Louis Archinard pour glorifier son expédition ? consisterait à trouver le juste équilibre avant toute décision entre ce qui est moral aujourd'hui, ce qui était légal hier et ce qui répond à l'impératif permanent de contextualisation historique. concerne la légalité, il y a matière à discussion puisqu'une grande partie des collections venues d'Afrique, exposées aujourd'hui dans nos musées, répond parfaitement à la légalité de l'époque.

Comment éclairer le politique, sur lequel repose aujourd'hui le processus de restitution, afin d'éviter qu'il ne s'apparente au fait du prince ? Comment faire en sorte que le ministère de la culture et les conservateurs jouent pleinement leur rôle dans ce processus pour éviter que des atteintes fondamentales ne puissent être portées aux principes mêmes qui sont au coeur de notre politique muséale ? car aujourd'hui ce sont les propositions du rapport Sarr-Savoy qui font foi pour nos interlocuteurs. C'est sur ses inventaires, en dépit de leurs inexactitudes, qu'ils s'appuient pour formuler leurs requêtes. Si le dernier mot doit revenir au politique, cela ne doit être qu'en vertu d'une décision éclairée par des avis étayés et non pour répondre à je ne sais quelle tyrannie de l'instant, aux seules raisons d'une diplomatie du ou pour donner des gages à telle ou telle approche mémorielle, pour ne pas dire communautaire. Ce serait jeter par-dessus bord les principes multiséculaires forgés précisément pour que le patrimoine de la Nation ne soit jamais soumis aux humeurs du prince de l'instant. sage précepte scellé sous le règne de Charles IX, sur l'initiative du chancelier Michel de L'Hospital. Il est certes difficile d'élaborer une loi-cadre posant des critères précis qui ne soient ni trop larges, au risque d'être contraires à la Constitution, ni trop rigides, au risque d'empêcher des restitutions qui paraîtraient opportunes. Des solutions permettant de protéger l'inaliénabilité des collections publiques et la vision universaliste de nos musées, tout en ne fermant pas la porte à un dialogue des cultures, doivent pourtant être trouvées au plus vite, car le risque est grand que nous ne soyons de plus en plus fréquemment bousculés par des demandes de plus en plus nombreuses. Or votre projet de loi n'esquisse aucune doctrine en matière de transferts de biens culturels, de circulation des collections et de leur monstration au public.

Il se limite à l'exécution d'une décision présidentielle. Il n'en provoque pas moins un réel et profond malaise j'évoquerai la manière de procéder des auteurs du rapport Sarr-Savoy, qui n'ont pas jugé bon d'auditionner la présidente de la commission de la culture du Sénat, alors qu'ils ont pris le temps de rencontrer son homologue de l'Assemblée nationale. Permettez-moi donc de douter de la qualité de leur démarche, très certainement militante et assurément

renforcé par la mise en extinction de la Commission scientifique nationale des collections, chère à Philippe Richert et à Catherine Morin-Desailly. Notre pays avait pourtant là l'outil pour s'emparer du sujet et y réfléchir de manière scientifique. Hélas, rien n'a été fait pour faciliter le travail de cette commission. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui à nous retrouver dans une position défensive. davantage quand vous nous dites que le caractère inaliénable des collections est maintenu. Mais, madame la ministre, cette loi d'exception étant fondée, sinon sur le fait du prince, du moins sur la raison d'État, elle en appellera d'autres au rythme des demandes qui vont se multiplier La loi n'est pas encore votée que le président du Bénin, Patrice Talon, se dit « insatisfait ». Déjà cinq pays africains frappent à la porte et demandent le retour de 13 000 objets.

non seulement à ces artistes, mais à ces Africains ou ces Européens qui se sont battus pour sauvegarder ces oeuvres, c'est de tout faire pour qu'elles reviennent. » Votre projet de loi sera donc suivi d'autres, et comporte un risque sérieux d'atteinte à la cohérence des collections de nos musées, constituées au fil des siècles, et par là même à leur vision universaliste, fondée sur la mise en valeur du génie humain, d'où qu'il vienne. madame la ministre, je crois primordial d'ancrer à nouveau le caractère inaliénable de nos collections comme principe fondateur de l'universalité de nos musées, sauf à ouvrir la porte à un engrenage dont on ne sait où il s'arrêtera. Après tout, le retrait de la collection Dodds, général africain de l'armée française, n'est-il pas déjà une ? Dernière

pour ensuite les muséifier pour partie en Europe, mais aussi en Afrique. Je vous encourage donc, mes chers collègues, à adopter l'amendement que j'ai déposé avec Bruno Retailleau pour changer l'intitulé de cette proposition de loi en l'expurgeant du mot « restitution », qui sous-entend que notre pays aurait à expier je ne sais quelle faute morale. Mes chers collègues, j'entends bien la demande des pays africains, je ne la conteste pas. Mais je suis profondément mal à l'aise quant à la manière dont le Gouvernement entend y répondre, en cédant à une vision moralisatrice de notre histoire et en sacrifiant les principes qui participent de la grandeur de notre pays, au premier chef ceux de l'universalisme, fondateur même de notre conception de la citoyenneté. J'aurais tellement préféré que nous restions fidèles à l'héritage du président Jacques Chirac. Il était l'artisan infatigable d'une politique culturelle moins ethnocentrée, le fondateur du musée du quai Branly, dont la raison d'être, comme cela est inscrit dans sa charte, est le dialogue des cultures. Et s'il a offert le sceau du dey d'Alger au peuple algérien, c'est en le faisant acquérir par la France lors d'une vente aux enchères, et non en le faisant disparaître de nos collections nationales. Il est bien dommage que la France ne se soit pas dotée, dans son sillage, d'une vraie politique d'échanges et de circulation et d'une solide réflexion sur le sujet. Ce défaut de réflexion anticipée peut surprendre, tant la prégnance de la question est une évidence. Catherine Morin-Desailly nous a proposé, en commission, un amendement tendant à instaurer un conseil destiné à statuer sur les restitutions, une ébauche de régulation allant dans le bon sens. Elle esquisse une méthode, un cadre, une vision appelés par notre groupe. C'est la raison pour laquelle nous suivrons les préconisations de la rapporteure. Le groupe Les Républicains soutiendra ce projet de loi parce qu'il a été amendé en commission et que, désormais, il fixe pour l'avenir des procédures indispensables à la protection de nos collections et à l'universalité de nos musées. Nous voterons donc le texte issu de la commission, mais resterons très vigilants quant à la suite de la procédure parlementaire. Il y va de l'avenir de nos collections, de la préservation de notre patrimoine, de l'intégrité de notre histoire

vouloir restituer de façon temporaire ou définitive les oeuvres d'art africain des collections publiques françaises aux pays africains dont sont issues ces oeuvres. Dans cette perspective, il a confié à deux chercheurs, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, le soin de réaliser un rapport sur la restitution du patrimoine africain. Ce rapport se présente comme un plaidoyer en faveur d'une restitution massive, au nom de la repentance politique, du patrimoine africain présent dans les collections publiques françaises. Sont visées les oeuvres acquises « en l'absence de consentement des populations locales », par « la violence ou la ruse ou dans des conditions iniques ». Le rapport prévoit également la restitution des pièces saisies lors de conquêtes militaires, collectées lors de missions scientifiques ou par des agents de l'administration coloniale, ainsi que le retour des oeuvres issues du trafic illégal après 1960. La France détient près de 90 000 oeuvres d'art africain dans ses collections publiques, dont les deux tiers au sein des collections du musée du quai Branly. La remise du rapport au Président de la République, le 23 novembre 2018, a été l'occasion pour ce dernier d'annoncer la restitution de vingt-six oeuvres conservées actuellement au musée du quai Branly- statues de l'homme requin ou du roi Ghézo notamment -et réclamées depuis 2016 par la République du Bénin. Il s'agit du trésor de Béhanzin saisi comme butin de guerre en 1892, lors de la prise du palais d'Abomey par les troupes du général Dodds. De la même façon, le 17 novembre 2019, Édouard Philippe s'est engagé à restituer au Sénégal le sabre d'El Hadj Omar, fondateur de l'empire toucouleur et guide spirituel de la plus grande confrérie soufie du Sénégal, tiré des collections du musée de l'Armée, mais déjà confié au musée de Dakar pour une durée de cinq ans. Si le texte présenté replace sur le devant de la scène la difficile question de la restitution des oeuvres d'art africain, de nombreux conservateurs dénoncent la position manichéenne des auteurs du rapport susmentionné, arguant que « les musées ne doivent pas être otages de l'histoire douloureuse du colonialisme ». Ils s'alarment du préjudice pour les collections publiques, vitrine de l'art africain en Europe. Les risques liés à de mauvaises conditions de conservation sont bien réels, tout comme les risques de vol et de malversation dans des sociétés marquées par une forte corruption et une faible implication des autorités publiques dans les politiques patrimoniales. L'artiste Romuald Hazoumè dénonçait en 2016 une « culture béninoise à l'abandon », le délabrement des musées de son pays, les nombreux vols subis. Il qualifiait la restitution du trésor royal de fausse bonne idée, dans la mesure où le pays n'aurait pas les moyens ni la volonté de protéger et valoriser ces oeuvres. À l'image du grand sabre sacré, volé en 2001 au sein même du palais royal d'Abomey, les vols, incendies et l'absence de qualification du personnel rendent les conditions d'accueil des oeuvres actuellement conservées au musée du quai Branly difficiles. Le financement d'une autre structure, le musée de l'épopée des amazones et des rois du Dahomey, par un prêt de 12 millions d'euros de l'AFD devrait permettre de remédier à ce problème. Pour autant,

Il apparaît légitime de favoriser l'accès au patrimoine historique et culturel de la jeunesse africaine, source d'inspiration pour la création et de compréhension de son héritage culturel. loi, le groupe Les Indépendants considère aussi que de nouvelles formes de partenariat sont à imaginer. De nombreuses combinaisons sont possibles en matière d'engagements mutuels sur la formation des conservateurs, ou encore sur la valorisation et la protection d'oeuvres d'art qui, bien qu'issues d'un pays, d'une région, d'un peuple, représentent une richesse culturelle au rayonnement plus vaste, à la résonance internationale, qui appartient à l'humanité dans son ensemble. Les musées du monde entier témoignent de l'universalité de l'art, dont le propre est bien de dépasser les langues, les civilisations, les frontières, et de rapprocher les peuples.

le Bénin et le Sénégal, des biens culturels appartenant pleinement à leur histoire. Le trésor de Béhanzin, nommé d'après Béhanzin I, dernier roi du Dahomey, présente le dernier ensemble de pièces régaliennes de l'empire désormais disparu. Saisi en 1892 et rapporté en France par le général Alfred Amédée Dodds, ce trésor est un symbole important pour le Bénin, un vestige ultime d'une aire d'indépendance et de prospérité. Le sabre d'Omar Seydou Tall, dit El Hadj Omar, est nommé d'après le nom de son propriétaire. Chef spirituel soufi, érudit musulman et fondateur de l'empire toucouleur, ce dernier régna sur des territoires situés aujourd'hui au Sénégal, en Guinée et au Mali, vers les années 1850.

Ces deux objets sont donc des prises de guerre, des biens acquis dans la violence d'une époque de conquêtes coloniales qu'il nous faut aujourd'hui regarder avec lucidité. Les demandes de restitution du Bénin et du Sénégal sont donc tout à fait légitimes, et c'est en se fondant sur cette légitimité que le Gouvernement nous propose ce projet de loi. Celui-ci fait également écho à un engagement du Président de la République, pris le 28 novembre 2017 devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, et qui a suscité de grands espoirs au sein de la jeunesse africaine. Affirmons-le ici sans détour, notre groupe est favorable à ces restitutions, qui sont des témoignages de l'humanisme devant animer notre politique de coopération culturelle. En revanche, nous estimons qu'il faut sortir aujourd'hui de la logique de ces lois d'exception, obligeant le législateur à examiner chaque restitution dans un texte spécifique. Cette législation au cas par cas s'explique, bien entendu, par le principe d'inaliénabilité, lequel affirme que les biens appartenant aux collections publiques françaises ne peuvent être vendus ou cédés, mais elle freine cette amorce de politique de coopération culturelle volontariste. Les écologistes sont évidemment attachés au caractère inaliénable des collections publiques, qui garantit l'unité du patrimoine culturel au bénéfice de toute la Nation.

pour sortir de cette politique d'exception permanente, dont personne ne peut se satisfaire. Malheureusement, cet amendement ne sera pas examiné, ayant été déclaré irrecevable. Nous estimons toutefois que nous ne pourrons nous affranchir de cette réflexion essentielle. le Bénin et le Sénégal ne seront pas les seuls pays à avoir des demandes légitimes. Mali, Cameroun, Nigeria, Éthiopie, Tchad : plusieurs pays ont déjà fait des demandes, portant parfois sur des milliers d'objets ou de biens. Avec une politique de coopération culturelle enrichie d'un cadre législatif pérenne, nous pourrons durablement regarder notre passé en face, avec honnêteté, et renforcer nos liens avec de nombreux pays. Il s'agit non pas de repentance, mais simplement de justice

Madame la ministre, mes chers collègues, le groupe écologiste votera ce projet de loi, qui va dans le bon sens, tout en appelant à une réflexion plus globale sur l'évolution de notre législation, pour plus d'efficacité et de justice dans notre politique de coopération culturelle. La parole

ce projet de loi prévoit le retour au Bénin, leur terre d'origine, de vingt-six objets du palais de Béhanzin conservés au musée du quai Branly et la restitution au Sénégal d'un sabre et de son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, chef toucouleur. Il fait suite à une demande expresse de ces deux États. Il ne met pas fin au caractère inaliénable de nos collections publiques. Il témoigne d'une exigence de vérité, d'un souhait commun d'apaiser des conflits de mémoire, d'une confiance en un partenariat équilibré. Il faut se réjouir de cette coopération ! Ce projet de loi concrétise un engagement fort du Président de la République, prononcé en novembre 2017 devant les étudiants de l'université de Ouagadougou. Plus de la moitié de la population africaine a aujourd'hui moins de 25 ans. Dans mon département d'outre-mer, entre côtes africaines et Madagascar, la croissance de la démographie est sept fois plus forte que la moyenne nationale et les moins de 18 ans sont majoritaires. C'est une grande chance, mais aussi un lourd défi, pour Mayotte comme pour l'Afrique. Et nous savons l'importance, pour la construction harmonieuse de tous ces jeunes, de la connaissance de leur propre histoire. Peu de jeunes Sénégalais ou Béninois ont les moyens de voyager, de venir en France pour voir ces objets. Les restitutions-

-leur permettront d'accéder chez eux à des oeuvres de leur culture, de leur civilisation et de se les approprier. Ces oeuvres ont une forte portée symbolique. Apportées en France lors de l'expansion coloniale comme des objets de curiosité exotique, elles avaient d'abord, pour la plupart, une fonction spirituelle. Témoins d'un passé prospère, elles participent à un sentiment de fierté, de confiance en soi de populations trop souvent dépouillées de leur histoire. Il est donc important qu'elles soient exposées à tous- le Bénin et le Sénégal s'y sont engagés -et présentent des garanties de bonne conservation, dans le cadre d'une coopération repensée. La réalisation concrète du nouveau musée d'Abomey s'inscrira dans cette vision. Ces biens, revenus à leur terre originelle, ne seront certes plus notre propriété, mais ils resteront toujours porteurs d'universel, parce qu'issus du génie humain. Nous restons vraiment, avec ce texte, dans le domaine de l'exception. C'est pourquoi la création d'un comité chargé d'émettre un décidée par notre commission, ne me semble pas opportune. Nos musées nationaux resteront, avec leurs collections, des vecteurs de connaissance de l'autre et d'histoire partagée. Prêts et expositions temporaires doivent se multiplier afin de profiter au plus grand nombre. Certes, on peut croire que des demandes de restitution, limitées jusqu'à présent, se feront plus nombreuses et pourront sembler tout aussi légitimes. Mais ce sera à la France de décider, au cas par cas, en fonction d'ailleurs des terres de conflits, hélas propices aux destructions et aux pillages.

Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants votera ce projet de loi. La parole

madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit ce jour vise à sortir des collections nationales vingt-sept biens culturels, afin d'ouvrir la voie à leur restitution à deux pays africains, le Bénin et le Sénégal.

le sabre, attribué à El Hadj Omar Tall, inscrit à l'inventaire des collections du musée de l'Armée, officiellement réclamé par le Sénégal depuis juillet 2019 et exposé au musée des civilisations noires de Dakar depuis son inauguration en décembre 2018, dans le cadre d'une convention de dépôt entre la France et le Sénégal. L'ensemble de ces oeuvres constitue des prises de guerre. Les vingt-six objets béninois, issus du palais des rois d'Abomey, ont été emportés en 1892 par le général Dodds, commandant des armées coloniales françaises, dans le cadre de la guerre du Dahomey qui l'opposait au roi Béhanzin. Le sabre attribué à El Hadj Omar Tall aurait, quant à lui, été confisqué à Ahmadou Tall, son fils, par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893. est une nouvelle étape au sein d'une réflexion de plus grande ampleur : d'une part, celle du Président de la République, Emmanuel Macron, relative au patrimoine africain présent en France et, d'autre part, celle qui est liée à l'universalisme culturel, voulant que les oeuvres culturelles appartiennent, au-delà des frontières des pays d'origine ou d'accueil, au patrimoine de l'humanité.

Le retour de ces objets tend à atteindre un double objectif : le premier est de permettre à la jeunesse, mais aussi à l'ensemble de la population africaine d'avoir accès en Afrique à son propre patrimoine le second est de consolider le partenariat, ici dans sa dimension culturelle, entre la France et le continent africain- il s'agit donc d'un objectif diplomatique et de coopération. Le groupe Union Centriste est favorable à ces motifs, mais cet accord de fond ne doit pas occulter les réserves sur la forme et la méthode que nous souhaitons émettre. fait que notre intervention ici, en tant que législateurs, est aujourd'hui moins démocratiquement souhaitée que juridiquement requise. Les objets concernés sont des prises de guerre, non des biens volés. Ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de la convention de l'Unesco de 1970. Dès lors, c'est le droit français qui s'applique. un principe prévaut : celui de l'inaliénabilité des collections publiques, consacré par la loi et s'opposant à ce que la propriété d'un bien conservé dans les collections publiques puisse être transférée. Le législateur doit donc intervenir pour poser des exceptions : c'est la raison de ce texte. Le principe de la restitution des oeuvres béninoises a été acté par le Président de la République en novembre 2018. Le sabre, lui, a d'ores et déjà été restitué au Sénégal, le prêt n'étant qu'une sorte d'étape transitoire « en attendant » que le Parlement français ne valide la décision gouvernementale. Ainsi, ce projet de loi entérine une décision présidentielle, alors même que le principe législatif d'inaliénabilité est inscrit dans la loi pour éviter dans ce domaine le « fait du prince », même si, ici, je le souligne, les raisons sont tout à fait acceptables. On demande au Parlement de consacrer en droit ce qui est d'ores et déjà acté en fait. Ce n'est pas cela le rôle du Parlement ! La deuxième réserve que le groupe Union Centriste souhaite émettre s'inscrit dans une réflexion plus générale, qui aurait dû et doit être engagée à propos de ce patrimoine. Lors de l'examen en 2009 de la proposition de loi, déposée par ma collègue Catherine Morin-Desailly, visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections, le ministre de la culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, s'était exprimé en ces termes au sujet de l'initiative parlementaire : « Elle Elle marque surtout l'ouverture, trop longtemps retardée à mes yeux, d'un véritable débat de fond sur le recours au déclassement, en donnant aux collectivités publiques les moyens de disposer en la matière d'une doctrine définie en parfaite concertation. » Tout est dit Plus d'une décennie et deux mandatures présidentielles plus tard, d'aucuns pourront constater que ce véritable débat de fond sur la nécessité d'établir une doctrine a malheureusement peu avancé. malheureusement », parce que, citant de nouveau le ministre en 2009, « la question qui nous est posée à l'occasion de l'examen de la présente proposition de loi est de celles qui attisent la controverse, les prises de position morales ». Cela aurait effectivement mérité que les gouvernements s'en saisissent C'est précisément pour éviter controverses et procès que la Commission scientifique nationale des collections a été créée en 2010. Elle devait permettre à la France d'engager une réflexion prospective. Faute pour le ministère d'avoir donné à cet organe les moyens de réussir, la France se trouve désormais dans une démarche sujette à la critique, défensive et casuistique. Coup de grâce, la loi d'accélération En l'absence de doctrine et de critères au sujet du retour des oeuvres, nous sommes en effet contraints de n'avancer que par lois spécifiques portant exception au principe d'inaliénabilité. Eu égard aux dizaines de milliers d'oeuvres qui sont et seront réclamées par les États, et dans une démarche proactive que commande la restitution de biens mal acquis, nous ne pouvons raisonnablement pas considérer que les lois d'exception itératives soient satisfaisantes. Madame la rapporteure a donc justement, et nous l'en remercions, présenté à la commission un amendement visant à créer un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d'oeuvres d'art extra-occidentales. Il aura pour objectif d'apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision en la matière d'encourager notre pays et, en particulier, le monde muséal à approfondir sa réflexion sur ces questions qui ont vocation à rebondir dans les années à venir, afin de ne pas prendre les décisions au fur et à mesure, et d'anticiper ; de contenir dans le futur le risque de décisions conjoncturelles, aussi versatiles que l'actualité et l'opinion de l'instant ou les orientations politiques du moment. Enfin, ce conseil est tout à fait indispensable pour poser une doctrine en matière de retour et contenir ce risque de « fait du prince », non seulement par principe, mais aussi pour les conséquences que cela emporte pour les oeuvres. On ne restitue ni ne conserve : il doit y avoir une décision objective, qui s'appuie sur une argumentation posée et construite. L'enjeu du débat autour des restitutions consiste à concilier ce qui était légal autrefois avec ce qui est moral aujourd'hui, pour reprendre les mots de ma collègue Catherine Morin-Desailly. Prendre du recul, exprimer la ou les vérités, voilà les raisons pour lesquelles il faut que le conseil proposé par la rapporteure soit mis en place, avec les moyens de fonctionner. Son travail permettra de concilier la portée universaliste de nos musées avec les exigences tout à fait légitimes des pays africains, comme c'est ici le cas. Nos histoires sont mêlées et communes, chargées d'un héritage parfois lourd, mais rien n'est manichéen, et le danger serait de résumer ce parcours de l'humanité à un simplisme caricatural. Ces oeuvres ont une charge morale forte et symbolique, mais elles sont le témoin de la complexité de la construction de notre monde et de la place majeure qu'occupe la culture dans la construction de l'humanité. La culture de l'autre est un bien commun, notre bien commun. La culture de l'autre a changé notre culture. Le groupe Union Centriste votera donc en faveur du texte, avec une vigilance accrue quant aux efforts réalisés par le Gouvernement pour qu'une doctrine sur la question des restitutions soit discutée et établie.

séminaire de recherche « Parcours d'objets » organisé par la Direction générale des patrimoines et l'Institut national d'histoire de l'art, le renforcement des équipes au musée du quai Branly-Jacques Chirac grâce à des bourses de recherche spécifiques et un poste de recherche.

ne peut conduire à la restitution ou au don des oeuvres. Il ne peut pas y avoir de doctrine plus claire et plus affirmée ! Toute autre procédure viendrait la battre en brèche et serait

je n'éprouve pas pour autant les craintes que semblent traduire certains propos, mettant en doute les capacités des peuples africains à assurer la conservation de ces oeuvres.

tend à supprimer l'article 3, ajouté par le Sénat, qui crée un conseil national de réflexion sur la circulation et le retour d'oeuvres d'art extra-occidentales.

de ces objets et que vous comptiez le prolonger. D'ailleurs, pour avoir également eu des échanges avec des représentants du ministère des affaires étrangères, j'ai cru comprendre que, sur cette question, un travail interministériel se dessinait pour l'avenir.

modèle Montmorency, 1820, fabriqué en Haute-Alsace -, il a été donné par un général français et repris par un général français ! Est-ce vraiment ce qu'aurait choisi le Sénégal ?

Où va-t-on s'arrêter ? L'an dernier, le Parlement belge a voté une résolution tendant à engager un dialogue

le choix des oeuvres doit obéir aussi à une logique culturelle et patrimoniale. Vous avez fait remarquer, à juste titre,

approprié d'élargir le périmètre du conseil national à l'ensemble des cas extra-européens, plutôt qu'extra-occidentaux, afin de lui permettre de se prononcer sur les demandes qui pourraient émaner d'autres pays eux eux aussi précédemment colonisés : je pense à l'Amérique du Nord, à l'Australie ou encore à la Nouvelle-Zélande- je suis bien placée pour le dire. En revanche, pour ne pas alourdir excessivement l'appellation du conseil,

mon ministère, s'appuyant sur l'avis des spécialistes des musées concernés, conserve une préférence pour la première formule, comme le montrent les journées professionnelles et les séminaires de recherche qu'il organise, avec des musées nationaux

: loi de 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud et loi de 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories

d'en avoir précisé l'esprit est d'avoir confirmé que le mot « restitution » comporte bien une charge morale. Je rappelle qu'un examen attentif de ce qui était légal dans le contexte de l'époque disqualifie

il ne s'agit pas de nier l'histoire telle qu'elle s'est passée, seulement de reconnaître une juste part de responsabilité. Il convient non pas de regarder l'histoire d'hier avec les yeux d'aujourd'hui, mais de légiférer pour aujourd'hui et demain.

L'universalisme que nous invoquons depuis le début de cette discussion nous oblige à rendre accessibles ces biens culturels à l'ensemble des pays qui nous les demandent, et pas seulement à ceux qui ont les moyens financiers de les accueillir. Ce devoir est d'autant plus impérieux quand il s'agit de les offrir à la contemplation des sociétés qui les ont réalisés et que nous en avons privées. Je regrette vivement que ce débat ait été enfermé dans les limites juridiques étroites d'un texte consistant en des transferts de propriété. Il eût été utile de nous interroger sur la validité, presque morale, d'un acte de propriété sur des oeuvres qui n'ont cessé de passer de main en main et de traverser les frontières et les époques. Pour reprendre l'exemple des chevaux de Saint-Marc, que valent les droits de leurs derniers propriétaires, alors qu'ils témoignent aussi du génie grec, de la capacité de la Renaissance constantinienne à fonder un nouvel empire sur les bases de l'Antiquité finissante et, finalement, du lien jeté entre l'Orient et l'Occident par la République de Venise ? Les oeuvres qui nous intéressent ce soir ont été juridiquement incorporées dans les collections nationales françaises, ce qui justifie notre débat sur ce texte. Néanmoins, elles participent surtout de l'expression du génie humain. À ce titre, la France n'en est que l'ultime dépositaire ce statut lui donne sans doute des droits, mais lui confère aussi des devoirs envers celles et ceux qui n'y ont pas accès, en particulier les populations auxquelles nous les avons arrachées. Si notre pays continue de défendre l'universalisme du patrimoine mondial et des musées, il ne peut continuer à opposer cette conception aux légitimes demandes de partage. Nous devons abandonner cette position strictement défensive et nous engager dans une politique qui favorise les échanges et la circulation de toutes les oeuvres